des données aux fins de recherche et de développement. Le groupe CRCE y est opposé. Même si le Gouvernement assure que les données conservées et exploitées à des fins de recherche et développement ont vocation à être anonymisées, et que, ainsi, cette mesure n'aura aucun impact sur les particuliers, nous n'en avons aucune certitude. D'ailleurs, cet article n'en apporte pas la garantie. Comme le note La Quadrature du Net, prenant l'exemple de la, la NSA, et des sociétés privées comme Palantir, l'article 8 autorise la conservation jusqu'à cinq de toutes les informations obtenues dans le cadre d'opérations de renseignement. En théorie, les informations ainsi conservées ne pourront plus être exploitées qu'à des fins de recherche et de développement d'outils de renseignements divers.

En l'occurrence, le Conseil d'État pointe le risque d'un « détournement à des fins de surveillance » des données, si celles-ci ne sont pas « matériellement et informatiquement cloisonnées

Ainsi, un mois après le recueil, les services de renseignement sont contraints de supprimer l'audio et de garder certaines vidéos qui sont muettes, ce qui les rend difficilement exploitables. Pour échapper à cet écueil, l'Assemblée nationale a harmonisé, en première lecture, les durées maximales de conservation en les alignant sur la durée la plus élevée, soit cent Or, comme le précise la délégation parlementaire au renseignement, la DPR, dans son dernier rapport, « l'augmentation de trente à cent vingt jours de la durée de conservation des enregistrements sonores, [ ...] serait, de l'avis de la délégation, susceptible d'être jugée

Par conséquent, le présent amendement tend à réduire la durée de conservation proposée par l'Assemblée nationale pour cette technique de renseignement spécifique, sans préjudice de l'alignement des durées de conservation qui répond à une difficulté rencontrée par les services. En outre, cette nouvelle durée, plus raisonnable, permettrait d'éviter une censure du Conseil constitutionnel.

l'efficacité. Outre la question de la conservation des données, le principe même de la validation de la conservation massive de données à des fins de recherche et de développement pose des difficultés sur le fond. C'est d'autant plus vrai que le mécanisme de contrôle prévu paraît largement insuffisant. La CNCTR dispose uniquement de la possibilité d'adresser une recommandation au Premier ministre tendant à la suspension d'un programme de recherche, lorsqu'elle estime qu'il ne respecte plus les conditions posées dans le texte. Mais à ce moment du processus, le mal sera déjà fait. Voilà pourquoi nous estimons que ce dispositif doit faire l'objet d'un encadrement dans la durée et que le Parlement doit se saisir de nouveau du sujet à l'extinction de cette période expérimentale. Quel

instaure un régime autonome de conservation des renseignements pour les besoins de la recherche et du développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements.

pose problème. Tout d'abord, il est impossible de garantir un cloisonnement parfait des données informatiques, lesquelles, du fait de leur exposition, pourront toujours faire l'objet d'un piratage.

des techniques de collecte, d'extraction et de transcription mises en oeuvre par les services, afin que la CNCTR soit en capacité d'exercer pleinement le contrôle sur la durée de conservation de tels renseignements, cette durée pouvant aller jusqu'à cinq ans après leur recueil. À cette fin, il paraît nécessaire, en l'absence de décret d'application, de prévoir un registre faisant apparaître la date de recueil pour assurer leur destruction en tout état de cause à l'échéance fixée par l'article 8 du projet de loi. Ce type de registre me semble également utile dans le cadre de la collecte des renseignements et de leur exploitation bien comprise. Quel est l'avis de

qui, sans mésestimer les garanties prévues à l'article 8 du projet de loi, préconise de prévoir des précautions supplémentaires lorsque les programmes de recherche et de développement portent sur des techniques mises en oeuvre au moyen d'un traitement algorithmique. Quel est l'avis de

par l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que la CNCTR émet un avis sur la demande d'autorisation relative au traitement automatisé et sur les paramètres de détection retenus. L'avis est défavorable.

des fins de recherche et développement. Nous souhaitons que les données n'ayant aucun lien avec une quelconque menace terroriste ne puissent pas être utilisées au-delà d'une durée de deux ans. années proposé par le Gouvernement apparaît bien trop long lorsque les informations ne permettent pas d'identifier les signaux faibles d'une éventuelle menace terroriste. Nous proposons donc que ces données ne soient plus utilisées deux ans après leur recueil et

indispensables à la validation des capacités techniques de recueil et d'exploitation, sous le contrôle de la CNCTR. Une durée de deux ans nous paraît trop courte pour faire de la recherche et du développement sur des techniques complexes.

des données, ne permettrait pas d'atteindre l'objectif du texte et réduirait très fortement la capacité des services à développer des outils d'enquête pertinents. Par ailleurs,

le comprend bien, il s'agit d'installer partout sur le territoire des antennes factices permettant de recueillir la totalité des données de connexion des usagers de téléphonie mobile. Le projet de loi vise à adapter cette technique de captation générale des informations à la nouvelle technologie de la 5G, dans laquelle les identifiants des terminaux deviennent temporaires. on constate que ce que d'aucuns nous présentent comme un progrès vous contraint à transformer vos techniques de renseignement. Ce n'est donc sans doute pas un progrès pour tout le monde

pour intercepter le trafic des communications mobiles, récupérer des informations à distance ou pister les mouvements des terminaux. Son utilisation inquiète les défenseurs de la vie privée, car ce dispositif n'est pas conçu pour les écoutes ciblées.

contre le terrorisme : « Il ne faudrait pas que les technologies prévues pour intercepter les communications d'individus que l'on a intérêt à surveiller permettent, du même coup, d'écouter d'autres personnes qui ne devraient pas l'être. » Si cette technique est pour l'instant réservée à certaines procédures judiciaires concernant des infractions graves à la loi pénale, elle risque d'entraîner une surveillance de masse du fait de la récolte de renseignements qui ne sont pas liés à une menace terroriste. Elle est donc particulièrement attentatoire aux libertés et à la vie privée des personnes. La CNIL s'était d'ailleurs inquiétée de son utilisation,

résultat. L'article 10 autorise simplement la réquisition des opérateurs, notamment par les services de renseignement et par les services d'enquêtes judiciaires,

D'une part, l'expérimentation de cette nouvelle technique risque de conduire au recueil d'informations qui ne concernent ni la mesure ni la prévention d'actes terroristes, compte tenu du champ d'interception des communications rendu possible.

de la vie privée des personnes qui ne sont pas visées par la recherche de renseignements. Nous ne sommes pas forcément opposés à une expérimentation de cette technique

D'autre part, il apparaît évident que cette expérimentation, comme toutes les autres avant elle en matière de renseignement et de sécurité intérieure, finira par être pérennisée.

sont faites : augmentation des pouvoirs de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, contrôle des échanges avec les services étrangers, réel pouvoir de contrôle parlementaire, véritable possibilité de contestation individuelle. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à supprimer cet article. Quel

Sur le fond, cette restriction n'apparaît pas souhaitable, et ce pour deux raisons. D'une part, limiter la technique aux seuls services du premier cercle apparaît contradictoire avec l'objectif même de la modification législative envisagée, qui consiste non pas à ajouter un nouvel outil à l'arsenal des services de renseignement, mais uniquement à combler le déficit opérationnel qui pourrait résulter du changement technologique induit par l'émergence des terminaux de communications satellitaires. Les services appartenant au second cercle de renseignement sont également susceptibles de subir les conséquences néfastes du déport de certaines communications vers les moyens satellitaires. Il est donc indispensable que leur soit également ouverte la possibilité de recourir à cette technique. Cela ne fera pas obstacle à ce que, dans la pratique, pour des questions à la fois de coût et de technique, la mise en oeuvre effective des interceptions soit effectuée par les services du premier cercle, pour le compte des services du second cercle. D'autre part, d'un point de vue constitutionnel, le seul fait que le service demandeur de la mise en oeuvre d'une telle technique soit un service du second cercle

toute façon accéder à une interception de sécurité classique pour les finalités considérées. Par ailleurs, sa demande est soumise à l'avis de la CNCTR et est autorisée par le Premier ministre.

Le présent amendement vise donc à réintroduire la possibilité de désigner les services de renseignement du second cercle comme bénéficiaires potentiels de cette nouvelle technique de recueil de renseignements.

: La parole est à M. Jean-Yves Leconte. Par cet amendement, nous souhaitons apporter une précision utile sur le champ de l'expérimentation d'une technique qui est encore en voie de développement. L'article 11 autorise, à titre expérimental, les services de renseignement à intercepter, par le biais d'un appareil ou d'un dispositif technique, des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire, lorsque des raisons pratiques ou de confidentialité font obstacle au concours des opérateurs. Ce type de technique de renseignement est susceptible de permettre la collecte systématique et automatique de données concernant des personnes pouvant n'avoir aucun lien autre qu'une proximité géographique avec la personne visée par les services. Certes, l'article 11 précise que les correspondances interceptées seront détruites en l'absence de lien apparent avec la cible recherchée. Néanmoins, il subsiste le lien géographique. convient donc de circonscrire précisément la nature de ce lien, afin de permettre à la CNCTR d'assurer un contrôle effectif, si nécessaire, lorsqu'elle sera amenée à accéder aux opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées. Quel est l'avis de

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires émet un certain nombre de réserves sur cette nouvelle technique, notamment parce qu'elle risque de conduire au recueil d'informations n'ayant pas

Prenant acte de l'avis rendu par le Conseil d'État, les auteurs de cet amendement estiment que, sans enrichissement de l'étude d'impact sur ce point de la part du Gouvernement, l'expérimentation ne saurait aller au-delà au-delà du prochain renouvellement de la majorité parlementaire, qui, le cas échéant, pourra de nouveau se prononcer sur son maintien. Quel

Les mois passent, les années parfois, et aucun rapport ne nous est remis par le Gouvernement. Cet amendement vise donc à renforcer le pouvoir de contrôle parlementaire s'agissant de l'évaluation des résultats de l'expérimentation prévue au présent article. Afin de pallier le problème précité de non-transmission des rapports prévus dans la loi en matière de renseignement, le groupe Écologiste - Solidarité et et Territoires propose de mettre en place une obligation d'adresser au Parlement un rapport d'étape avant l'échéance des mesures prévues par le présent article. En En l'absence de transmission de ce rapport, l'expérimentation serait automatiquement suspendue et ne pourrait reprendre qu'une fois le rapport transmis au Parlement.

afin précisément d'éclairer le législateur. Ce délai de six mois permettra d'apprécier les résultats de l'expérimentation au plus proche de son échéance et mettra ainsi le Gouvernement en mesure de donner au Parlement une vision la plus complète possible, avant qu'il ne soit amené à se prononcer sur une éventuelle pérennisation de la technique. Par ailleurs, j'indique que, au-delà de la remise d'un rapport, le Parlement, notamment sa délégation au renseignement, dispose de prérogatives de contrôle qui lui permettront, s'il le souhaite, d'interroger le Gouvernement sur la mise en oeuvre de cette technique, sans attendre l'issue de l'expérimentation. L'article 17 du projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission des lois permet à ce titre à la DPR d'assurer le suivi des enjeux d'actualité et des défis futurs qui se rapportent à la politique publique du renseignement.

mais nous sommes au regret de constater l'absence d'évaluation précise et détaillée de ces mesures : aucun chiffre, aucun bilan, positif ou négatif, de l'utilisation des algorithmes contenus dans ces « boîtes noires » ne nous a été communiqué. Ainsi, le rôle du Parlement est une nouvelle fois entravé.

La CNIL le rappelle, une telle technique porte une atteinte particulièrement forte à la vie privée des individus et au droit à la protection des données à caractère personnel. Elle dénonce le caractère généralisé, à l'ensemble de la population, de cette pratique. Par ailleurs, de tels dispositifs sont techniquement les biais de conception des algorithmes ont des effets pervers relevés par les experts et bien documentés. Enfin, en l'état, l'étude d'impact ne permet pas de conclure à la nécessité de pérenniser le Conseil d'État le relève également -, car elle comporte très peu d'indications sur la mesure de l'efficacité opérationnelle de la technique couverte par le secret de la défense nationale.

Les journalistes et les chercheurs pourraient être les premiers à modifier leur mode de travail, afin de ne pas faire l'objet d'une surveillance.

Il joue donc un rôle indispensable, en raison de la nature même de l'évolution de la menace terroriste. En effet, celle-ci est de plus en plus endogène, elle se développe en marge des réseaux terroristes structurés, à distance et par voie numérique ; elle est par conséquent très difficile à détecter. Isoler certaines signatures électroniques sur internet constitue donc un complément naturel du travail ciblé sur les groupes, les réseaux et les individus terroristes, mais aussi du travail de renseignement humain conduit par nos services. Ce travail est central, mais il ne permet pas de tout couvrir.

Le taux d'alerte est donc très mesuré. Non, les services ne surveillent pas en masse ; non, ils ne sont pas noyés sous les alertes.

Ces derniers doivent obtenir l'autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR, pour lever l'anonymat des données issues d'une alerte. Enfin, le projet de loi prévoit de nouvelles garanties, dont la destruction immédiate de toute donnée non nécessaire, ainsi que la limitation aux services du premier cercle. La suppression de ces algorithmes conduirait à se priver volontairement d'un système efficace,

imaginez, mes chers collègues, que, à la suite d'une élection, notamment présidentielle, ce ne soit plus le cas ; imaginez qu'un gouvernement, moins favorable aux libertés individuelles, se saisisse de cette technique pour faire un fichage complet de la population Il faut donc réellement faire attention à ce que nous faisons, parce que nous pouvons donner des outils extrêmement dangereux de contrôle de la population à des gouvernements qui auraient des intentions moins légitimes que les vôtres, madame la ministre. La parole est à Mme Esther Benbassa,

l'extension des données traitées par les algorithmes, qui jusqu'ici ne concernaient que les données de trafic et de connexion de téléphonie, aux adresses complètes internet met en place un domaine nouveau d'investigation, plus attentatoire à la protection de la vie privée et des données personnelles. » Plus généralement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires exprime des craintes sur les risques de surveillance généralisée de la population et déplore que le législateur soit tenu d'inscrire définitivement un tel dispositif dans un projet de loi sans disposer d'évaluation précise dans une étude d'impact. Quel

Les individus que les algorithmes visent à détecter utilisent massivement les moyens de communication électroniques et ils utilisent beaucoup plus internet que la téléphonie classique. Même les individus peu formés aux techniques clandestines savent qu'il est beaucoup plus sûr d'utiliser les applications chiffrées sur internet que leur forfait téléphonique classique. Il ne m'est pas possible de vous détailler les utilisations dans lesquelles ces URL sont nécessaires sans compromettre nos algorithmes, mais je peux néanmoins prendre un exemple qui me paraît très parlant

Cette propagande se trouve aujourd'hui sur des sites de plus en plus clandestins, du fait de la lutte qui est exercée contre la diffusion de tels didacticiels. Un algorithme fondé en partie » -sur la consultation ou sur le téléchargement de ces vidéos est envisageable et démontre l'intérêt de disposer de ce type de données.

Les services de renseignement n'ont accès à aucune de ces données. La CNCTR contrôle l'architecture et les paramètres des algorithmes proposés, leur fonctionnement et leurs résultats et elle intervient à chaque étape du processus en cas de renouvellement de l'algorithme, lors d'une demande de levée d'anonymat d'une donnée qui a produit une alerte ou même dans le cadre de son droit permanent d'accès à toute information, comme aux locaux des services. Le texte renforce encore ces garanties en réduisant au strict nécessaire la durée de conservation des données et en limitant au premier cercle le maniement de cette technique,

Le recueil des URL pourrait porter atteinte à la vie privée des personnes, en ce qu'il pourrait faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances d'ordre privé ; cela a été dit. Il n'est aucunement démontré que cette surveillance accrue des Français constitue un moyen efficace de lutte contre le terrorisme, qui est l'objet principal du présent projet de loi. En aucun cas le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne saurait accepter une telle disposition. C'est pourquoi il demande la suppression de cet alinéa.

Il est donc tout à fait inutile de prévoir que les URL figurant dans le contenu des correspondances électroniques ne puissent être traitées par l'algorithme. Cela laisserait

à l'ensemble des URL, les traitements algorithmiques prévus à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Le présent amendement a pour objet de supprimer ce caractère expérimental, qui est inutile à plusieurs titres. la technique de l'algorithme a d'ores et déjà donné lieu à une expérimentation, qui a été prolongée à plusieurs reprises. Nous disposons désormais du recul suffisant et de tous les enseignements utiles pour perfectionner cet outil. le rappelle, les algorithmes sont indispensables pour la détection de la menace terroriste, nous en avons parlé ; plusieurs États européens y ont recours. L'efficacité de ces outils sera d'autant plus grande que ceux-ci pourront concrètement traiter, au-delà des seules données téléphoniques, les données internet. Je l'ai indiqué, je le répète, chacun le sait, c'est par internet que passe aujourd'hui l'essentiel des communications. La loi permet déjà, en principe, de traiter les données internet, mais, en pratique, les algorithmes ne peuvent pas distinguer entre les URL qui sont de pures données de connexion et celles qui sont des données mixtes, c'est-à-dire qui révèlent indirectement une partie du contenu de la communication.

Nous renforçons encore substantiellement les garanties qui entourent la mise en oeuvre de l'algorithme. Seul un nombre très résiduel de données peut, finalement, être transmis aux services de renseignement, uniquement à ceux du premier cercle et à l'issue d'une procédure très contrôlée faisant intervenir plusieurs autorisations du Premier ministre, qui ne peuvent elles-mêmes être exécutées qu'avec l'accord

au plus tard le 31 juillet 2024 sur le sujet spécifique de l'extension à toutes les URL. Il appartiendra alors aux membres du Parlement d'en tirer les conséquences en prenant les initiatives, y compris législatives, qu'il jugera appropriées. En matière de lutte contre le terrorisme, le Parlement doit doter les services de renseignement des outils efficaces, c'est-à-dire proportionnés et stables, qui permettent une action dans la durée. est l'objectif du présent amendement que vous propose le Gouvernement, éclairé par l'expérimentation des quatre années qui s'achèvent.

ne serait-ce que pour assurer la conformité du dispositif au droit constitutionnel et au droit européen. Par ailleurs, le faible niveau de développement des algorithmes- autant que nous puissions en juger -incite à prévoir une expérimentation et un nouveau rendez-vous

et susceptibles d'être recueillies par les services de renseignement « ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications ». De ce fait, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires

du 21 avril 2021. Nous considérons sa rédaction largement en deçà du cadre fixé par le Conseil d'État. En effet, cet article ne modifie qu'à la marge le système existant, qui oblige les opérateurs à conserver pendant un an l'ensemble des données de connexion des populations, alors que ce système a été jugé en grande partie

Cet article instaure une surveillance de masse, autorisée à titre exceptionnel, mais qui sera systématisée en pratique. Ainsi, sur injonction du Premier ministre, l'ensemble des opérateurs internet et de téléphonie auront l'obligation de conserver pendant un an les données de connexion généralisées et indifférenciées d'une partie de la population. Ces mesures de surveillance sont disproportionnées, car elles autorisent le placement sous surveillance de vastes franges de la population pour des motifs très larges et imprécis, et ce sans aucun contrôle judiciaire. La conservation généralisée et indifférenciée de certaines données de trafic et de localisation peut être imposée sur injonction du Premier ministre, pour une durée maximale d'un an, renouvelable à l'issue d'un réexamen de l'état des menaces pesant sur la sécurité nationale. Seul est prévu un recours devant le Conseil d'État, après Seul est prévu un recours devant le Conseil d'État, après l'injonction. En tout état de cause, cette mesure fait l'objet d'un contrôle insuffisant et viole les obligations fixées par la Cour de justice de l'Union européenne, qui exige, dans son arrêt du 21 décembre 2016, le contrôle du juge en amont ou d'une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande par conséquent la suppression de cet article.

mais ce ne sera probablement pas suffisant. Il est possible qu'un certain nombre d'enquêtes soient fragilisées par le manque de robustesse des dispositions telles qu'elles sont proposées par le Gouvernement. Il me semble que le droit européen, lorsqu'il pose problème à de nombreux États européens, doit être changé.

ne pourront plus recourir à des réquisitions de données de connexion dans le cadre d'enquêtes liées à la criminalité ordinaire. En effet, le dispositif mis en place par l'article 15 se limite à la criminalité grave. C'est la raison pour laquelle il nous a paru important de mieux

il faut accepter d'aller plus loin ensemble. Je ne pense pas que l'article 15 soit réellement la panacée, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux en l'état actuel du droit européen. Ce dernier n'est pas un droit divin ; on peut le modifier si on le souhaite. Nombreux sont nos partenaires européens

Le Conseil d'État avait par ailleurs exigé, dans son arrêt du 21 avril 2021, un contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir d'avis conforme ou par une juridiction. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu, le 25 mai, un arrêt, dans lequel elle exige que les activités d'interception en masse soient soumises à l'autorisation d'une autorité indépendante dès le départ, dès la définition de l'objet et de l'étendue de l'opération.

et celui du Conseil d'État du 21 avril 2021 allaient tous deux dans le sens d'un contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir d'avis

a été dit précédemment, en cas d'urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné la mise en oeuvre immédiate de la technique autorisée, il est possible de passer outre le caractère suspensif de la saisine du Conseil

Il s'agit ici de mettre notre droit interne en conformité avec l'arrêt de la CJUE précité, qui permet la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion autres que les adresses IP « aux seules fins de sauvegarde de la sécurité nationale lorsqu'un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, sur injonction d'une autorité publique, soumise à un contrôle effectif d'une juridiction ou d'une autorité administrative indépendante

Le présent amendement tend à mettre en place un droit d'information des personnes concernées par les mesures prévues à l'article 16. En effet, quand une personne fait l'objet de mesures de surveillance, elle n'est pas avertie lorsqu'il y est mis fin. L'objectif du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est donc de renforcer le droit d'information en matière de surveillance, car nous estimons qu'il est tout à fait normal

: La parole est à M. Jean-Yves Leconte. Nous sommes favorables au principe de l'article 16, qui vient renforcer le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur le territoire national, en conférant un caractère contraignant à ses avis, tout en ménageant une exception en cas d'urgence. il nous paraît nécessaire d'articuler strictement les prérogatives constitutionnelles de l'exécutif et les pouvoirs de contrôle dont est dotée la CNCTR- autorité administrative indépendante -, combinés avec le recours éventuel au Conseil d'État en cas de désaccord avec le Premier ministre. Le recours à la procédure d'urgence soulève des interrogations légitimes, en particulier au regard de l'existence d'un réel contrôle. Nous avons bien conscience qu'il n'est pas possible de limiter les conditions dans lesquelles l'urgence pourrait être invoquée par le Premier ministre ou de lui imposer un avis conforme en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, s'agissant en outre d'une matière relevant de la police administrative. Il importe néanmoins de rappeler que, en tout état de cause, dans l'hypothèse où le Conseil d'État, saisi par la CNCTR, jugerait que la technique de renseignement a été mise en oeuvre sans urgence suffisamment caractérisée, il pourra, en application de l'article L. 773-7 du code de justice administrative, annuler l'autorisation délivrée par le Premier ministre et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Nous proposons donc, par cet amendement, de rappeler que la procédure prévue à l'article 16

Elle propose ainsi d'être informée des recommandations adressées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à l'exécutif tendant à l'interruption de la mise en oeuvre d'une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés en cas d'irrégularité constatée. est effectivement essentiel pour la DPR de disposer, chaque année, d'un bilan des recommandations adressées par l'autorité administrative indépendante, et ce afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en oeuvre ou exploitées en méconnaissance du code de la sécurité intérieure.

Il s'agira essentiellement de préciser les services, les techniques de renseignement et les finalités concernés par lesdites recommandations. Pour rappel, les membres de la délégation, de même que les fonctionnaires composant son secrétariat, sont habilités au niveau « secret-défense

au renseignement et à renforcer ses prérogatives. La délégation parlementaire au renseignement n'est actuellement composée que de quatre députés et quatre sénateurs, dont les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité intérieure et de défense, qui en sont membres de droit. Par le présent amendement, nous souhaitons donc renforcer son effectif et le porter de huit à vingt membres, afin d'accroître le pluralisme politique de cet organe et et de permettre la représentation des groupes minoritaires et de l'opposition. Pour gagner en effectivité, la délégation parlementaire au renseignement doit également disposer d'un pouvoir d'injonction renforcé

dans les faits, d'une représentation. Il nous paraît donc impératif d'étendre la composition de la délégation parlementaire au renseignement, d'une part, pour renforcer le caractère démocratique de cet organe et, d'autre part, pour gagner en effectivité du contrôle. Quel est l'avis de

Pour répondre aux exigences de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État, dans sa décision du 21 avril 2021, a imposé au Gouvernement de procéder, sous le contrôle du juge administratif, un réexamen périodique de l'existence d'une menace pour la sécurité nationale afin de justifier la conservation généralisée des données de connexion imposée aux opérateurs par le droit français. Voilà six ans, le Parlement avait prévu une disposition permettant à la délégation parlementaire au renseignement d'auditionner, chaque semestre, le Premier ministre sur l'application des dispositions de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. En première lecture, curieusement, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Il serait néanmoins utile de la remplacer par une audition annuelle du Premier ministre sur le réexamen périodique de l'état de la menace, qui sous-tend le maintien de la conservation généralisée des données de connexion, comme l'exigent la CJUE et le Conseil d'État. en effet, qu'un contrôle parlementaire puisse s'exercer sur le sujet et que l'exécutif motive sa position. À ce titre, il est proposé que la délégation parlementaire au renseignement,

Nous souhaitons que, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les moyens affectés au renseignement humain, en particulier à l'échelon territorial, et sur les formations dispensées aux agents de renseignement.

Or leur rôle est aussi de travailler au plus près de la population, pour prévenir et lutter contre les crimes, les délits, mais aussi toute forme de radicalisation, en récupérant les renseignements à la source et en collaborant avec nos services de renseignement. est à Mme Esther Benbassa. Au moment où le Gouvernement souhaite faire de la surveillance technologique une priorité en misant sur des moyens numériques de surveillance et de collecte de données, il est important de valoriser le renseignement humain. Aujourd'hui, nous observons une nette progression des nouvelles technologies, avec la montée en puissance de métiers liés à la cybersécurité, la surveillance des télécommunications, la cyber-infiltration ou encore la mise en oeuvre d'anonymisation les crypto-monnaies. Pourtant, selon un article du de 58 des 59 attentats déjoués entre 2013 et 2019 l'ont été grâce au renseignement humain. Si, à l'ère numérique, le rôle des nouvelles technologies au service de la lutte antiterroriste est important, ces dernières ne doivent pas justifier l'extension de la surveillance de masse. Certes, les outils de surveillance apportent une aide au renseignement français, mais l'intervention humaine est décisive et c'est elle

des antennes du renseignement territorial et des cellules de renseignement départementales, nous ne disposons actuellement, en tant que parlementaires, d'aucune information précise sur les moyens affectés au renseignement humain et à la lutte antiterroriste. Cet amendement vise à rappeler l'importance capitale du renseignement humain à l'échelon territorial pour déjouer les projets d'attentat.

de loi prévoit la création d'une base légale permettant l'usage de dispositifs de brouillage afin de lutter contre les drones malveillants qui pourraient constituer une menace contre les personnes ou les biens, « pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales

(dont des centrales nucléaires ou des prisons) constatés chaque année et de l'utilisation connue de drones sur les théâtres d'opérations extérieures, il est nécessaire de se doter d'un cadre légal permettant l'usage de dispositifs de brouillage par les services de l'État. » Cet article pose également la question de l'étendue des brouillages. Le Commissariat aux communications électroniques de défense et l'Agence nationale des fréquences s'en assureront

Dès lors, une fois la loi promulguée, il appartiendra au service d'archive d'identifier les documents. De plus, tous les services publics d'archive disposent aujourd'hui- ce n'était pas le cas en 2008 -de systèmes d'information archivistiques permettant une gestion optimale, car automatisée, de la collecte et de la communication des documents. Par ailleurs, les administrations des archives ont d'ores et déjà entrepris, parallèlement à nos travaux parlementaires en cours, des repérages permettant d'identifier, notamment par le biais de leur description ou de l'identité de leurs producteurs, les fonds d'archives dont les critères de communicabilité seront susceptibles d'être modifiés par le présent texte. Enfin,

a rappelé que seul le délai de cinquante ans est constitutionnel et que toute restriction à ce délai pose un grave problème. La seule manière d'apporter

des archives publiques ! Comme l'ont affirmé mes collègues, les associations de chercheurs, d'historiens et les services publics d'archives s'émeuvent du nouveau dispositif

de faciliter le travail de ces personnes, qui contribuent à notre mémoire collective, en sanctuarisant l'accès aux archives publiques. Et voilà que la majorité sénatoriale et le Gouvernement ne souhaitent pas aller dans ce sens ! Étant moi-même chercheuse et historienne, je ne peux que le regretter. Le privilège des démocraties, c'est de laisser leurs historiens écrire le passé, en regardant le présent.

le principe de base est celui de la libre communicabilité des archives publiques. Dès lors, ces restrictions ne font pas du tout honneur à notre pays, à la recherche et à la science Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la rédaction actuelle de cet article. Nous regrettons, une fois de plus, que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ne s'interrogent pas sur leur positionnement

permet un équilibre substantiel entre le code du patrimoine et le code pénal- on voit bien aujourd'hui qu'un conflit existe entre ces deux textes.

L'article 19 fixe le régime juridique de la communicabilité applicable aux archives intéressant la défense nationale, en posant comme principe que « toute mesure de classification [ ...] prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit ».

Bien entendu, nous comprenons l'impératif lié à la défense nationale dans la mesure où les documents concernés sont d'une particulière sensibilité et où leur communication prématurée pourrait être de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation. Toutefois, le dispositif retenu ne propose pas les garanties attendues permettant aux archivistes, aux historiens, aux chercheurs et aux universitaires d'être en mesure d'exercer leur métier, au service de la mémoire collective.

cet amendement vise à prévoir que la prolongation de la durée d'incommunicabilité doit avoir un caractère exceptionnel et être justifiée par une menace grave pour la sécurité nationale en cas de divulgation des documents.

profondément la loi de 2008, en inversant l'ordre des facteurs ! Si nous ne définissons pas de manière précise les critères susceptibles d'appeler une prolongation du délai

Les archives du monde d'hier permettent de comprendre celui d'aujourd'hui et de bâtir celui de demain. En la matière, notre Constitution est claire. L'article XV de la Déclaration des droits de l'homme proclame : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Le législateur a posé un principe simple : les archives sont communicables de plein droit au bout de cinquante ans, hormis les plus sensibles, notamment celles qui sont liées au nucléaire. Or ce consensus a été récemment remis en cause, tout d'abord par l'instruction générale interministérielle 1300, qui a contraint à une déclassification, c'est-à-dire à une décision administrative, avant que les archives ne deviennent

effet, justifier la présence d'un article qui limite autant l'accès à des pans importants de notre histoire collective, dans un texte ayant pour objectif de lutter contre le terrorisme ? Cet amendement est le fruit d'une discussion avec des historiens non seulement respectueux des principes constitutionnels et de l'esprit des lois de 1979 mais aussi soucieux de protéger les intérêts fondamentaux de l'État. Il est le reflet d'une position d'équilibre transpartisane et consensuelle.

quelques années. Le présent amendement vise expressément à prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa du délai. Ce recours permettrait

relatif au régime de communicabilité des archives classifiées. En effet, pour désigner les services de renseignement du second cercle, l'alinéa 9 de l'article renvoie aux « services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés par décret en Conseil d'État ».

Nous pensons que ce n'est pas pertinent, car c'est trop restrictif. La protection doit s'appliquer aussi à des documents qui permettent à la France d'avoir un avantage stratégique sur d'autres pays ; je pense notamment aux études réalisées sur des techniques.

à l'échéance de ce délai. En outre, le fait qu'un tampon de déclassification n'ait pas été apposé sur le document ne sera plus un obstacle.

elle ne ménage pas une conciliation équilibrée entre le droit d'accès aux archives et la nécessité constitutionnelle de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. ? Dans certains cas très particuliers, l'expiration du délai de cinquante ans ne met pas fin à la sensibilité des documents et donc à la nécessité de différer leur communication.

Je ne prétends pas que toute la communauté des historiens y souscrit. Je vous demande simplement d'entendre qu'un large panel d'historiens y a participé

Il a fallu mettre au point un système légal permettant de concilier ces différents objectifs. C'est dans cette perspective que nous avons essayé d'identifier, en les circonscrivant au mieux, quatre nouvelles catégories de documents pour lesquelles il n'est pas possible de fixer par avance un délai au-delà duquel toute sensibilité aurait disparu.

Tout d'abord, la prolongation de la durée d'incommunicabilité restera exceptionnelle : ce qui le garantit, c'est le caractère ciblé et résiduel des catégories de documents pour lesquelles une prolongation sera possible.

le document deviendra communicable à l'instant même où il perdra sa sensibilité. Ainsi, pour ce qui concerne les armes ou les équipements, c'est tous les ans que le Gouvernement actualisera la liste des documents accessibles

aux documents dont la divulgation représenterait une menace grave pour la sécurité nationale. Sur ce point aussi, je vais m'efforcer de vous assurer. Le Conseil d'État n'a émis aucun doute sur la constitutionnalité de ces dispositions ; si certains commentateurs ont cru déceler des opinions contraires dans les conclusions prononcées voilà deux semaines au contentieux, devant le Conseil d'État, je peux vous affirmer

Quant aux documents qui restent détenus par les services qui les ont produits et qui sont également des archives publiques, ils n'ont vraisemblablement jamais fait l'objet d'un quelconque inventaire. Cela signifie qu'il faudra rechercher, puis passer en revue l'ensemble des documents susceptibles de bénéficier d'une prolongation à l'issue du délai de cinquante ans.

Par ailleurs, contrairement à ce que vous avancez, le rapporteur public du Conseil d'État a clairement indiqué que, selon lui, il n'y avait pas de primauté du code pénal sur le code du patrimoine. en l'état, la loi de 2008 est satisfaisante et que vos services peuvent protéger la sécurité nationale sur la base des principes constitutionnels.

Aux États-Unis, ces documents sont librement consultables après un certain délai ; ensuite, c'est aux administrations d'indiquer aux chercheurs et aux lecteurs ce qui est communicable de plein droit et ce qui ne l'est pas. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas adopter le même système,

Madame la ministre, vous nous appelez à traiter ce sujet avec sérieux : c'est ce que nous faisons,

votre point de vue. Vous avez cité trois associations avec lesquelles vous avez mené une concertation : l'association des archivistes français, l'association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'association Josette-et-Maurice-Audin. J'ai sous les yeux le communiqué de presse que ces trois associations ont publié le 28 juin dernier,

qui est consacré aux archives. L'enjeu est considérable. C'est une fermeture sans précédent de l'accès aux archives publiques qui se dessine avec l'article 19. » Deuxièmement, « contrairement à ce que soutient la direction des affaires juridiques du ministère des armées, l'immense majorité des historiens et des archivistes ne considèrent pas que le texte arrive à un bon équilibre ; ils pensent le contraire. » Troisièmement, « nous le disons donc sans détour : nous sommes très inquiets des effets pratiques de ce texte et plus largement de ce qui se joue avec ce projet de loi. et enfin, « les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d'État doivent permettre d'amender le texte afin d'éviter que la loi ne soit la première loi de fermeture des archives de l'histoire et que ne soit créé un régime dérogatoire au droit commun pour les services de renseignement. » C'est exactement dans ce sens que nous vous proposons d'amender le présent texte ! Ainsi, l'immense majorité des historiens et des archivistes

Les rédacteurs de ce projet de loi invoquent la valeur opérationnelle des archives du monde du renseignement.

Peut-on, aujourd'hui, écrire une histoire des mouvements de la Résistance en France durant la Seconde Guerre mondiale sans consulter les archives des services secrets de la France libre ? C'est difficile ! Pourtant, le Président français Emmanuel Macron avait annoncé vouloir faciliter l'accès aux archives, après la remise du rapport de l'historien français Benjamin Stora consacré aux questions mémorielles portant sur

ce mécanisme de déclassification automatique des documents d'archives publiques à l'expiration des délais prévus dans le code du patrimoine, quand on ne fait que revenir, par là, au texte de 2008. Autrement dit, on ne fait que mettre fin à des pratiques administratives

Le scrutin est clos.

Le scrutin est clos.

la décision du tribunal administratif ! Nous proposons donc quelque chose de simple et pratique : que, dans ce genre de cas, le juge compétent puisse ordonner, y compris en référé,

Même avis : défavorable.

qu'il faut traiter les causes et non les symptômes des crimes odieux commis au nom de l'islamisme politique, qui alimente la peur et attise la haine de l'autre pour propager les idéologies obscurantistes les plus mortifères, nous sommes convaincus, pour part, que notre État de droit doit être renforcé. Nous avons soulevé un certain nombre de questions, sur lesquelles je ne reviens pas, mais force est de constater que nous n'avons pas pas obtenu de réponses. Votre refus obstiné de débattre sur des sujets d'importance capitale pour notre sécurité, mais aussi

dans notre État de droit et respecte notre loi fondamentale, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain saisira le Conseil constitutionnel lorsque ce projet de loi aura été définitivement adopté par le Parlement.

Par ailleurs, les propositions constructives de la commission des lois en matière de suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme ont enrichi le texte qui sera adopté par le Sénat ce soir. À cette occasion, nous regrettons que le Gouvernement ait maintenu ses positions au sujet des Micas et nous déplorons les risques constitutionnels relatifs à la possibilité d'allonger leur durée à deux ans. En ce qui concerne la conservation des données de connexion sollicitées dans le cadre des enquêtes judiciaires, il nous semblait absolument nécessaire de ne pas les cantonner aux aux seuls faits de criminalité grave, au risque de mettre en péril nombre d'enquêtes menées au quotidien par nos policiers et nos gendarmes. Le texte qui sera voté par le Sénat ce soir renforce les moyens des services de lutte contre les nouvelles menaces, tout en apportant des garanties supplémentaires. Enfin, le dispositif adopté à l'instant à l'article 19 en matière d'archives publiques, sur proposition de Mme Canayer, nous semble concilier, dans la mesure du possible, protection du secret de la défense nationale et liberté de travail des chercheurs, historiens et archivistes. Je remercie chaleureusement les rapporteurs du travail de qualité qu'ils ont réalisé, malgré la complexité et la technicité particulières de ce texte.

regretter l'absence totale de concertation préalable. Je dénonce le recours à la procédure accélérée, dont le Gouvernement a pris l'habitude. Tous deux privent le Parlement d'un véritable débat. Je l'ai

Nous déplorons de nouveau le manque de cohérence entre les mesures existantes, ainsi que l'absence de réels moyens de prévention de la radicalisation, particulièrement en détention, particulièrement en détention, ce sujet n'étant jamais traité. Enfin, je tire la sonnette d'alarme, avec la Ligue des droits de l'homme : ce projet de loi confirme toutes les craintes exprimées depuis 2015 par plusieurs organisations de défense et de promotion des droits humains, ainsi que d'avocats et d'universitaires, en matière d'atteintes à l'État de droit

Le Gouvernement serait-il en train de perdre sa boussole s'agissant des principes de l'État de droit ? Notre groupe est fermement opposé à cette dérive sécuritaire prétendument justifiée par la lutte contre le terrorisme- une

dissimuler l'absentéisme des représentants de la Nation, s'il faut vraiment aller voter pour des absents. L'abstentionnisme a ses raisons, dirons-nous !

Personne ne demande plus à voter ? ... Le scrutin est clos.